La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale

avec une économie mondiale qui tourne au ralenti et des échanges commerciaux paralysés. La France doit se réapproprier son appareil de production ; c'est une nécessité vitale d'un point de vue alimentaire. Notre souveraineté alimentaire devrait être un objectif stratégique majeur. Vous nous direz, monsieur le ministre, sur le modèle de l'exception culturelle, cette exception agriculturelle permettrait de consacrer le principe suivant : notre modèle agricole et alimentaire ne saurait être appréhendé comme une simple marchandise soumise aux règles d'un marché hyperconcurrentiel

Pour autant, pratiquer l'exception agriculturelle, pour reprendre votre formule, mettrait en difficulté une grande partie de nos agriculteurs européens et français qui exportent. Je pense bien sûr aux viticulteurs, aux producteurs fromagers, aux céréaliers et aux planteurs de betteraves. faut évidemment que l'Europe muscle ses dispositifs pour ne pas avoir de déconvenues dans les négociations commerciales ; elle doit remettre la question de la souveraineté

Vous l'aurez compris, autant la commission est favorable à établir des échanges dans des conditions de concurrence loyale, autant elle ne pense pas qu'une exception agricole globale, telle que vous la proposez, soit opportune. Avis défavorable.

Cet amendement vise à réduire et à interdire progressivement l'usage des pesticides dans le secteur agricole. La contamination des aliments et de l'environnement par des résidus de pesticides pose un véritable problème en matière de santé publique et de protection de la biodiversité, s'agissant notamment de la capacité des écosystèmes à stocker du carbone. L'exposition chronique peut entraîner l'apparition de cancers, une perturbation du développement des foetus et des enfants et une perturbation des systèmes reproducteur, endocrinien et immunitaire. Malgré la prise de conscience accrue de la nocivité des produits phytosanitaires pour la santé humaine et le vivant, l'évolution des comportements reste beaucoup trop lente. Il convient de poursuivre les efforts dans ce domaine, en accélérant la diminution de l'usage des produits phytosanitaires dans le secteur agricole. Cet amendement s'inscrit dans une dynamique de réduction de l'usage de ces produits engagée par le Grenelle de l'environnement et le plan Écophyto. le nom de notre cher collègue Joël Labbé interdit depuis le 1 janvier 2017 l'utilisation des produits phytosanitaires par les personnes publiques dans les espaces verts, forêts et promenades ouverts au public et par les personnes privées dans leur jardin. Il convient désormais de s'attaquer à l'usage de ces produits dans le secteur agricole. Quel

; son expertise est reconnue. Ensuite, depuis 2008, deux plans Écophyto ont été mis en place afin de réduire progressivement l'utilisation de ces produits dans les zones agricoles et non agricoles. Je pense, pour ma part, qu'il faut privilégier cette logique d'accompagnement. Enfin, dernier point et non des moindres, quelle serait la conséquence d'une interdiction générale de l'usage de produits phytopharmaceutiques ? Concrètement, nous interdirions à nos agriculteurs de les utiliser alors que la plupart des denrées alimentaires que nous importons continueraient d'être élaborées avec ces produits.

L'amendement tend donc à ancrer le dispositif de certification de projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et de séquestration de carbone dans le secteur agricole afin de pouvoir valoriser économiquement

de séquestration de carbone dans le secteur agricole permettent de valoriser économiquement nos productions. Les exploitations pourront être accompagnées financièrement dans leur projet certifié label Bas-carbone grâce à des crédits carbone. Je suis donc favorable à cette précision que vous proposez. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Parmi ses nombreux objectifs- réduction des émissions de gaz à effet de serre, protection de la biodiversité, résilience des systèmes agricoles et alimentaires territoriaux -, il y a place pour une politique de l'alimentation durable. notre amendement vise à créer un lien de compatibilité entre les orientations fixées par cette stratégie nationale et celles qui sont définies dans les plans régionaux de l'agriculture durable. Notre objectif est d'assurer une cohérence entre la politique nationale et les politiques régionales en matière d'alimentation durable. Au niveau local, les projets alimentaires territoriaux (PAT) doivent d'ores et déjà répondre aux objectifs définis dans le plan régional

La rédaction de l'amendement n'a pas évolué, malgré la proposition qui vous avait été faite de prévoir, plutôt qu'un rapport contraignant de « compatibilité », pour reprendre les termes mêmes

est ainsi libellé : La parole est à M. Joël Labbé. Si la relocalisation de l'alimentation et la souveraineté alimentaire, très présentes dans la rédaction de l'article issu des travaux de la commission, sont des enjeux essentiels que nous soutenons, elles doivent aller de pair avec des objectifs forts sur le plan environnemental. Il nous est possible- c'est même nécessaire au vu de l'urgence écologique -de développer et de relocaliser notre production alimentaire tout en renforçant la performance écologique de notre agriculture et sa transition vers des modèles résilients et soutenables.

Cet amendement de repli vise à prévoir une nouvelle catégorie d'action dans le programme national pour l'alimentation : le rééquilibrage de la consommation de protéines végétales et animales. Afin de rendre la transition des élevages français et l'amélioration du bien-être animal économiquement viables, il convient notamment de consommer « mieux et moins » de viande, condition nécessaire pour limiter les importations de protéines animales de basse qualité

à l'article 61 et le programme national pour l'alimentation relèvent du niveau réglementaire. Ensuite, les ajouts que vous proposez d'insérer à l'alinéa 5 sont satisfaits par la mention de « l'empreinte carbone de l'alimentation », qui a été ajoutée en commission l'adoption d'un amendement que je défendais. donc pas nécessaire d'adjoindre encore de nouveaux éléments à cette énumération. Enfin, l'objectif que vous mentionnez d'un équilibre entre la consommation de protéines végétales et la consommation de protéines animales me semble en décalage avec la réalité de notre modèle agricole. nous ne sommes tout simplement pas en mesure d'assurer cet équilibre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Gouvernement a mis en place une stratégie nationale en faveur du développement des protéines végétales alors que, dans le même temps, en commission du développement durable, nous renforcions nos outils de lutte contre la déforestation importée afin de maîtriser l'empreinte carbone de notre alimentation.

Cet amendement vise à lier l'enjeu climatique du programme national relatif à la nutrition et à la santé, mis en avant dans ce texte, avec celui de la lutte contre la pauvreté. Une nourriture de qualité pour tous est un prérequis indispensable pour engager une véritable transition écologique. Cet amendement contribue à l'atteinte de l'objectif « moins de carbone, plus de justice ». Quel Cet amendement est satisfait par la mention de la « justice sociale », après laquelle vous proposez d'insérer « la lutte contre la pauvreté ». Cette précision n'est donc pas nécessaire ; elle pourrait même introduire une hiérarchie dans les objectifs, ce qui n'est pas souhaitable compte tenu de la rédaction actuelle de l'article. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

une vallée sinistrée par le manque d'eau. Cet amendement vise à favoriser l'installation de retenues collinaires.

terre d'élevage. Cela fait deux étés que les paysans passent leurs journées à rouler de l'eau et qu'on voit les vaches, au milieu de la route, chercher l'eau, quand elles ne crèvent pas de soif ; et on continue à leur dire : « Chers amis, il faut attendre ! » Nous vous demandons simplement des autorisations simples pour de

une démarche extrêmement importante. Je le redis, nous sommes disponibles pour travailler avec vous, à la place qui est la nôtre, et avec les partenaires professionnels concernés.

conformément aux recommandations de l'atelier 9 des États généraux de l'alimentation organisés en 2017. Actuellement, le schéma régional de santé comporte des volets consacrés à l'offre de soins et à l'accès aux soins, à la sensibilisation de la population et des professionnels aux maladies vectorielles ou encore à des besoins spécifiques liés à la situation géographique.

nous semble indispensable de rendre ce lien obligatoire, car déconnecter ces deux aspects ne nous semble pas en phase avec les études médicales, qui font de l'alimentation, au même titre que le manque d'activité physique, un élément déterminant dans l'apparition de certaines maladies. Cet amendement vise ainsi à ce que chaque schéma régional de santé intègre un volet consacré à l'alimentation.

C'est l'équivalent de 3,3 milliards de tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère, soit un peu moins de 10 % de notre empreinte carbone totale. Il s'agit d'un gaspillage de ressources naturelles autant qu'une cause notable de dérèglement du climat. La lutte contre le gaspillage alimentaire fait partie des axes structurants du programme national de l'alimentation et de la nutrition (PNAN) pour la période 2019-2023, réponse à la directive européenne n° 2018/851 engageant les États membres à réaliser un suivi du niveau de gaspillage alimentaire et à faire état des progrès réalisés. Cet amendement vise donc à attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de généraliser l'obligation de fournir des bilans chiffrés sur le gaspillage alimentaire. Quel

j'avais émis un avis défavorable, car l'article visé du code de la santé publique, qui est relatif au schéma régional de santé élaboré par l'ARS, comporte des objectifs de sécurité sanitaire et d'organisation des soins, mais ne mentionne pas d'objectif thématique de politique publique.

Cet amendement est donc satisfait dans l'esprit. Enfin, l'article 59 A, traité au fond par la commission des affaires économiques, prévoit que les formations continues et initiales relatives à la cuisine intègrent dans leurs référentiels des modules

Comme l'a démontré une récente note de l'Office français de la biodiversité (OFB), la certification environnementale est aujourd'hui un outil inopérant pour assurer la transition agroécologique et garantir la durabilité des produits agricoles, du fait des lacunes de son cahier des charges. L'OFB estime que « les seuils retenus ne permettent pas de sélectionner des exploitations particulièrement vertueuses ». Il critique ainsi la voie B d'accès à la certification : alors que le seuil maximal d'achat d'intrants y est fixé à 30

plutôt que de supprimer cet outil, qui doit permettre de valoriser économiquement nos producteurs. Ensuite, les objectifs de développement de l'agriculture biologique sont déjà pris en compte dans l'élaboration des PRAD, les plans régionaux de l'agriculture durable. Or, ainsi que nous l'avons prévu en commission avec plusieurs de mes collègues, également membres du groupe de travail « Alimentation durable et locale » commun à notre commission et à celle des affaires économiques, les projets alimentaires territoriaux seront compatibles avec les orientations fixées par les PRAD. Votre amendement est donc satisfait,

L'article 61 introduit à l'Assemblée nationale vise à permettre aux porteurs d'un projet alimentaire territorial d'engager une démarche collective de certification environnementale pour l'ensemble des exploitations agricoles contractantes. Cet article prévoit, en son alinéa 10, que, dans les espaces densément peuplés, ces projets participent prioritairement au renforcement de l'autonomie alimentaire locale et favorisent le développement de l'agriculture urbaine. Toutefois, la notion de priorité est inopportune en ce qu'elle limite la flexibilité offerte aux porteurs de projet dans l'élaboration des objectifs ; c'est la raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer toute référence à une priorisation des objectifs visés. En outre, l'alinéa 11 indique que, lorsqu'ils s'engagent dans la formalisation d'un projet alimentaire territorial, les gestionnaires des services de restauration collective favorisent la mise en oeuvre de projets communs sur un périmètre géographique, agricole et économique cohérent. Cette rédaction impose une obligation qui semble trop contraignante pour les PAT ; l'amendement a donc également pour objet de supprimer cette contrainte supplémentaire.

Les projets alimentaires territoriaux, parce qu'ils sont le vecteur d'une dynamique territoriale partagée et démocratique autour de l'alimentation durable et locale, sont des outils pertinents pour travailler sur le réemploi des contenants alimentaires. Il est ainsi proposé d'intégrer cette dimension complémentaire à la définition des projets alimentaires territoriaux. L'adoption de cet amendement contribuerait également à instaurer une transversalité et une cohérence entre les différents outils de développement local durable, garantes de l'efficacité de l'action publique. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement me semble aller un peu loin dans le détail des objectifs assignables aux projets alimentaires territoriaux, même si je partage bien sûr votre préoccupation,

dans le présent projet de loi sur l'initiative de ma collègue rapporteure Marta de Cidrac s'inscrivent dans la même logique et ont permis des avancées. En commission, nous avons ajouté d'autres objectifs, mais plutôt au niveau « macro », si vous me permettez l'expression.

monsieur le ministre,

Néanmoins, il convient d'aller plus loin, en prévoyant une couverture de l'ensemble du territoire en 2025. Les projets alimentaires territoriaux permettent de fédérer les différents acteurs d'un territoire autour de la question de l'alimentation, de construire des circuits alimentaires de proximité prenant en compte les dimensions sociale, environnementale, économique et de santé de ce territoire. En outre, ils rapprochent les citoyens consommateurs des producteurs.

Il s'agit aussi, par cet amendement, de permettre aux collectivités territoriales d'anticiper et de mieux se préparer à cet enjeu majeur, sans préjuger de l'échelle à laquelle les PAT sont définis, afin de conserver la flexibilité propre au dispositif.

même que l'ambition d'une réduction des émissions de peroxyde d'azote et d'ammoniac n'a de sens qu'à l'échelle européenne, au minimum. À notre seul niveau, la réduction serait minime et la seule conséquence serait de pénaliser nos agriculteurs

en raison du déplacement de la demande vers les engrais uréiques, dont le potentiel émissif en ammoniac est plus élevé que celui d'autres produits. C'est pourquoi un arrêté du 10 mai 2017 précisait qu'à partir de la campagne 2019-2020 l'autorisation de ce type d'engrais se ferait sous certaines conditions afin de limiter leur volatilisation. L'arrêté, signé par la ministre de l'environnement d'alors, prévoyait aussi qu'une étude serait mise en place en vue d'une taxation ou de la modulation de la fiscalité des engrais azotés. De fait, ce qui était proposé à l'article 62 issu de l'Assemblée nationale n'était autre qu'une traduction bien plus souple, concertée et échelonnée d'un dispositif conforme à nos engagements européens et, surtout, en phase avec l'urgence environnementale.

Il paie très cher des produits alimentaires- mais il y a des raisons objectives à cela : les coûts de production sont bien souvent plus élevés -et, par ses impôts, il paie les externalités négatives de certains autres types d'agriculture dont il ne consomme pas les produits. J'en appelle à plus de cohérence, à l'application du principe pollueur-payeur et à la prise en compte de toutes les externalités dans l'accompagnement des différentes agricultures. La parole

Privilégiant l'innovation sur l'injonction, l'engagement collectif sur la stigmatisation, nos commissions vous proposent, monsieur le ministre, la mise en place d'un plan d'accompagnement qui permettra d'atteindre les objectifs que vous avez établis en valorisant des solutions techniques qui existent, comme l'enfouissement ou la modification de certaines pratiques culturales.

N'envisageons la taxe qu'au niveau européen, afin de ne pas accabler encore les agriculteurs français. Cette position- vous le savez -est juste, pratique, opérationnelle ; elle permettra à la France de tenir ses engagements. Les

Alors que la Convention citoyenne pour le climat a pointé le poids important des engrais de synthèse dans les émissions de gaz à effet de serre, alors que l'étude d'impact du présent projet de loi reconnaît la taxation des engrais azotés comme une des mesures les plus nécessaires et les plus structurantes en la matière, le texte que nous examinons aujourd'hui est loin d'être à la hauteur des enjeux. En effet,

sans parler des risques et des accidents industriels, dont la fréquence et la dangerosité ont été rappelées dans un récent rapport commandé par votre gouvernement, monsieur le ministre, sur la gestion des risques liés à la présence d'ammonitrates dans les ports maritimes et fluviaux- c'est, là encore, un simple constat.

Ainsi le présent amendement tend-il à créer une redevance sur l'azote de synthèse. Je tiens à indiquer clairement, dès la présentation de cet amendement, qu'il ne s'agit pas d'une mesure visant à pénaliser les agriculteurs, mais plutôt d'une incitation à la transition agroécologique.

Les répercussions de l'usage des engrais azotés sur notre environnement, sur notre biodiversité, sur la santé de nos agriculteurs exigent une réponse forte telle que l'instauration de la présente redevance incitative. La réduction de l'utilisation des engrais azotés s'inscrit pleinement dans la transformation de notre agriculture vers un modèle raisonné et vertueux.

en concertation étroite avec la commission des affaires économiques et en lien avec la commission des finances. Les amendements n 1321 rectifié et 2035

Leur compétitivité-prix s'en trouvera donc dégradée, ce qu'ils ne pourront compenser par des hausses de prix, sauf à perdre les consommateurs français, en particulier les plus modestes. En contrepartie, les Français se tourneront vers des produits moins chers, donc souvent issus d'importations, ce qui ne participe pas à la maîtrise de l'empreinte carbone de notre alimentation. En outre, en l'absence d'alternative, les agriculteurs continueront à utiliser ces engrais. L'impact environnemental d'une telle mesure sera donc faible à court et à moyen terme. de ces contradictions, la commission a prévu la mise en place d'un plan d'accompagnement de la réduction de l'usage des engrais azotés, le plan Éco'Azot, sur le modèle de ce qui a été fait pour les produits phytopharmaceutiques.

avec le respect des objectifs de réduction des émissions de protoxyde d'azote et d'ammoniac, ce qui me paraît brutal. J'en viens à l'amendement n° 2177 du Gouvernement. Monsieur le ministre, je m'interroge. Le Sénat vous propose une voie de sortie par le haut

La fertilisation azotée est à l'origine de 42 % des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. Et pour cause ! Le surplus d'azote non consommé par la plante retourne dans l'atmosphère, principalement sous forme de protoxyde d'azote, dont le pouvoir de réchauffement est 298 fois- pas 300 fois, certes -supérieur à celui du CO2. Afin de respecter l'engagement de la France à parvenir à la neutralité carbone sur son territoire en 2050, les émissions de protoxyde d'azote

affectée au soutien des filières agricoles, notamment pour accompagner les investissements en faveur de la transition agroécologique. Monsieur le ministre, vous connaissez cet amendement : il vous a été présenté dans les mêmes termes à l'Assemblée nationale, par Dominique Potier. Je suis très curieux d'entendre l'avis de M. le rapporteur sur cet amendement de bon sens, qui vise

de contribuer à l'objectif de réduction de la fertilisation azotée minérale. Ainsi est-il proposé de supprimer la mention de « l'opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d'émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote des différents types d'engrais ». En effet, les émissions de protoxyde d'azote des engrais azotés étant très difficiles à différencier en fonction des produits et dépendant fortement de leurs conditions d'utilisation, cette solution n'est pas pertinente. Par ailleurs, nous proposons que le rapport étudie l'opportunité de des certificats d'économies d'engrais azotés, afin de ne pas faire peser sur les seuls agriculteurs les efforts de réduction de la fertilisation azotée minérale, mais aussi la possibilité d'établir une rémunération des pratiques vertueuses, en particulier par la mise en place de paiements que les modalités d'un renforcement de la formation, outil essentiel du changement des pratiques agricoles. Ces solutions semblent davantage susceptibles de garantir un véritable changement de pratique au sein des exploitations,

tend à revenir sur la position de la commission, qui a souhaité que le rapport prévu au second alinéa du II de l'article 62 étudie l'opportunité de fixer des taux de redevance différenciés en fonction des facteurs d'émission d'ammoniac et de protoxyde d'azote des différents types

Or la commission a supprimé cette mention, considérant qu'il s'agit d'un dispositif lourd sur le plan administratif, complexe à mettre en oeuvre et qui constituerait, là encore, une spécificité française, alors que la commission privilégie une approche européenne du sujet.

En effet, ce sont les surfertilisations qui ont le plus d'impact environnemental. Cette solution pourrait également constituer une alternative à la redevance, puisqu'elle ne crée pas de charge économique pour les agriculteurs, mais met en oeuvre une mesure garante d'une véritable réduction de la fertilisation. Elle devra être accompagnée de mesures fortes permettant aux agriculteurs d'assurer la transition de leur système de production.

fixer un objectif général pour l'ensemble du territoire national ne permet pas de prendre en compte les différences de fertilité des sols d'un territoire à l'autre. Dans certains cas, ce que vous proposez serait excessif ; dans d'autres, ce ne serait pas suffisant. Enfin, le plan Éco'Azot, évoqué à plusieurs reprises dans

Les articles 62 et 63 prévoient l'instauration d'un plan d'action national en vue de la réduction des usages d'engrais azotés, ainsi que la définition d'une trajectoire pluriannuelle de réduction des émissions de protoxyde d'azote et d'ammoniac du secteur agricole. Outre que le secteur non agricole ne faisait pas partie du champ initial du texte, la logique d'interdiction s'inscrit de manière frontale à rebours de la logique d'accompagnement adoptée par le Sénat lors de l'examen du texte en commission. C'est pourquoi, tout en conservant le principe d'une interdiction des engrais de synthèse à usage non agricole, le présent amendement vise à subordonner celle-ci à une évaluation préalable et à prévoir un délai d'adaptation suffisant pour permettre aux acteurs de s'y conformer.

néanmoins des standards de qualité nécessitant l'utilisation d'engrais de synthèse, par exemple les terrains d'entraînement. Ces terrains bénéficieraient ainsi d'une dérogation à l'interdiction prévue au présent article. L'amendement tend cependant à accompagner, pour ces espaces, la mise en place de bonnes pratiques environnementales de fertilisation, l'élaboration concertée d'une feuille de route. Enfin, cet amendement vise à clarifier la situation des hippodromes et des terrains d'entraînement de chevaux de course, pour s'assurer qu'ils entrent bien dans le périmètre de la dérogation.

la commercialisation et l'utilisation des engrais de synthèse pour l'entretien des espaces verts, hors vocation agricole. Certes, une dérogation est prévue pour les équipements sportifs, mais elle reste mal définie, car elle ne prend pas en compte les efforts que font les fédérations concernées, qu'il s'agisse du golf, des courses hippiques ou du football,

à ces nouvelles exigences réglementaires et s'oriente vers des engrais à libération lente ou progressive, comprenant parfois des biostimulants. Alors que nous sommes

Cet amendement vise ainsi à veiller à ce que la dérogation exonère les équipes sportives de l'interdiction d'utilisation d'engrais de synthèse.

C'est la raison pour laquelle nous avons voulu prendre en compte la situation des terrains de sport qui ne relèvent pas de la compétition officielle, mais dont les standards de qualité nécessitent l'utilisation d'engrais de synthèse, par exemple les terrains d'entraînement. En effet, pour ces terrains, l'utilisation de ces engrais est

qui a été déjà retenue à deux reprises dans la réglementation, dans le code général des impôts et dans celui de l'environnement. C'est une catégorie de référence pour le secteur des engrais non agricoles. cet amendement est issue des retours des professionnels du secteur. Il ne vise pas à changer le fond de l'article, mais à en clarifier la rédaction.

est ainsi libellé : La parole est à M. Joël Labbé. La mise en place d'une redevance sur les engrais azotés, accompagnée d'un surcroît de moyens et d'aides à la transition pour les agriculteurs, est essentielle. Afin de permettre au Parlement de se prononcer sur les moyens d'accompagnement et les modalités de mise en place de cette redevance

Nous disposons d'autres moyens pour suivre le respect de cette trajectoire, en lien avec l'article 62, tel qu'il a été réécrit par le Sénat : auditions de ministres ou de représentants des services d'administration, questionnaires ... La remise d'un tel rapport me paraîtrait un peu formelle. Nous aurons l'occasion de suivre la trajectoire mentionnée.

Ces dernières sont précisées dans les alinéas 4 à 6 de cet article. Or il est mentionné dans les cinq orientations de la SNDI que l'implication de l'État, couplée à l'action du secteur privé et des organisations de la société civile, est essentielle. La SNDI établit par ailleurs un dispositif de concertation, d'orientation et de suivi au sein du groupe national sur les forêts tropicales, afin de faciliter la mise en oeuvre de cette stratégie, son évaluation annuelle et ses révisions à venir. Par conséquent, il est inutile de mentionner dans la loi la composition des parties prenantes, ainsi que la plateforme déjà prévue dans la SNDI. L'objet de cet amendement

n° 1463, il me semble quelque peu prématuré. La plateforme de lutte contre la déforestation importée doit dans un premier temps permettre aux entreprises d'adapter leur chaîne logistique. Rendre ces données

pourrait encore évoquer le soja, l'huile de palme, ou les biocarburants, dont l'importation sera facilitée par la ratification du traité de libre-échange avec le Mercosur.

concerne également les produits ayant contribué indirectement à la déforestation, comme les biocarburants. En effet, elle couvre l'importation de matières premières ou de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation, à la dégradation des forêts, ou à la conversion d'écosystèmes naturels en dehors du territoire national.

l'objectif pour l'État de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation ou à la dégradation des écosystèmes. Pour l'heure, le champ de ce futur décret est très vague. Par notre amendement, nous proposons de le préciser davantage, car nous pensons qu'il est indispensable que ce décret traite

Sans traçabilité fiable, les opérateurs économiques ne pourront jamais savoir si leurs achats ne contribuent pas, d'une manière ou d'une autre, à la déforestation importée. La parole est à M.

qu'elles adoptent pour lutter contre la déforestation importée. Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, la France s'est engagée à soutenir et à renforcer ce dispositif. Or la liste des entreprises soumises au devoir de vigilance n'a toujours pas été établie.

de travail Alimentation durable et locale, que nous avons déjà évoqué. Contrairement à ce qu'écrivent les auteurs de l'amendement, le champ d'application de la loi sur le devoir de vigilance a été précisé par la rapporteure Marta de Cidrac à l'article 71 : il reprend désormais les préconisations d'un rapport d'inspection. La loi va donc gagner en effectivité, puisqu'elle s'appliquera aux grandes entreprises, au sens de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008. La suppression des seuils figurant dans le code de commerce constitue une vraie amélioration.

au plus près des réalités économiques, la lutte contre la déforestation importée et accompagner les entreprises dans la transformation de leurs chaînes d'approvisionnement. C'est aussi une exigence d'exemplarité qui est en jeu. La mise à jour de la liste ne me paraît pas, tant s'en faut, être une épreuve insurmontable : elle pourrait se faire tous les deux à trois ans. En tout cas, cette publication est une contrepartie à la précision du champ d'application de l'article 64 ,

engagée, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, à soutenir et à renforcer ce dispositif, la liste des entreprises soumises au devoir de vigilance n'est toujours pas

impliquerait une révision intégrale du PSN au moindre changement et rallongerait les procédures d'adaptation requises à chaque remise en cause, y compris pour des mesures très limitées et techniques.

En commission, Mme la rapporteure pour avis a indiqué que cet amendement était satisfait par les engagements pris par la France à l'échelon européen. Néanmoins, nous estimons nécessaire d'inscrire son dispositif dans la loi afin, justement, que personne n'oublie ces engagements à l'avenir. Pour rappel, le Pacte vert européen, ou, présenté en mai 2020 par la Commission européenne, vise à atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050 par la réalisation d'objectifs en matière de biodiversité et de préservation des ressources naturelles et des paysages.

en faveur de la biodiversité du Pacte vert européen. Il paraît à la fois cohérent et utile de garantir l'ambition du présent projet de loi en rendant le PSN compatible non seulement avec les stratégies nationales, mais aussi avec les stratégies prévues par le Pacte vert européen. La France doit s'engager pour le respect de ce dernier, d'autant qu'il est ambitieux pour la transition de notre agriculture comme pour celle de l'ensemble de l'agriculture européenne.

Merci

ou par des équipements appropriés. De plus, le système assurantiel actuel n'est pas rentable pour les assurances et ne peut être pérenne sans soutien public supplémentaire. Le renforcement du financement de ces acteurs privés, qui ont une vision comptable du secteur, ne peut toutefois être un objectif de politique publique s'il ne conduit pas à la protection effective des sinistrés à un coût raisonnable pour la collectivité. de 20 % de la surface agricole utilisée (SAU) française et mobilisent déjà considérablement les fonds publics, dont une part notable du budget du deuxième pilier de la PAC. De nombreux agriculteurs ne peuvent y avoir accès, soit du fait de tarifs inaccessibles, soit en raison de l'absence d'offres adaptées, par exemple en maraîchage diversifié. Ainsi, dans un contexte budgétaire contraint, toute nouvelle croissance des soutiens publics à l'assurance privée dans la PAC se fait nécessairement au détriment des autres objectifs du deuxième pilier et, notamment, de la transition agroécologique. Celle-ci contribue pourtant à la résilience des exploitations face aux aléas, notamment par la diversification des productions, l'autonomie des systèmes et le travail sur des variétés non-OGM résistantes au stress hydrique. À l'inverse, un système public financé par la PAC,

Afin de préserver un maillage agricole du territoire, il est nécessaire de soutenir les petites exploitations, qui permettent de bénéficier d'une production diverse et activité agricole dense. Le règlement de la prochaine PAC prévoit la possibilité de mettre en oeuvre un paiement forfaitaire pour les agriculteurs cultivant de très petites surfaces. Le renforcement du paiement redistributif serait une autre garantie de soutien aux petites exploitations ; il permettrait de restreindre les incitations à l'agrandissement des fermes et,, d'encourager le maillage du territoire par des exploitations agricoles nombreuses. Ces aides renforceraient en outre l'équilibre financier de petites exploitations, dans un contexte de fortes inégalités dans la distribution des aides de

au maintien de la biodiversité et des pollinisateurs. Il est important que cette agriculture soit reconnue

visent à la mise en place de systèmes de paiements pour services environnementaux (PSE), afin de rémunérer les externalités positives des pratiques vertueuses et d'inciter véritablement les exploitants à procéder

Mais il s'agit de PSE que l'on pourrait qualifier de « négatifs », à savoir de conditionnalités retranchant du revenu à ceux qui ne mettent pas en avant ces bonnes pratiques, à chaque fois que le budget de la PAC diminue. Ces PSE ne sont donc pas, à nos yeux, les bons véhicules pour aborder ces dispositifs.

chargé de suivre au plus près le déroulement du plan stratégique national.

avec la stratégie nationale bas-carbone (SNBC), la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB), le plan national santé environnement (PNSE) et la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI). Il s'agit là d'une proposition de la Convention citoyenne pour le climat.

aux produits issus du commerce équitable, définis par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, afin de rendre plus accessibles aux consommateurs des produits socialement et écologiquement responsables.

par la mise en oeuvre d'un plan d'action national au plus tard le 1 janvier 2022. Avec cet amendement, nous proposons d'aller plus loin en ajoutant aux objectifs de ce plan la juste répartition de la valeur au sein de la chaîne agroalimentaire. Il s'agit de mettre en lumière toutes les démarches novatrices qui ont vu le jour au cours des dernières années pour la production agricole et de reconnaître leur impact, aussi bien dans la lutte contre les inégalités que dans la valorisation économique de pratiques agroécologiques.

monsieur le ministre

qui vérifie la bonne articulation entre cette mesure nationale et le droit européen. Dès lors, la bonne application de la surtransposition est soumise à son accord. Dans les faits, cet accord est très difficile à obtenir et, même s'il est octroyé, il peut se révéler fragile : nous l'avons malheureusement constaté

les denrées alimentaires, notamment d'origine animale. Or une très grande partie de ces aliments proviennent de modes d'élevage allant à l'encontre de cette prise de conscience. C'est un constat : 97 % à 99 % des lapins sont élevés en cage ; 95 % des porcs sont élevés en bâtiments fermés sur caillebotis 85 % des poulets de chair sont élevés dans des hangars sans accès à l'extérieur ; enfin, plus de 50 % des poules pondeuses sont élevées en cage. Dans un souci de transparence, il nous semble nécessaire que les citoyens puissent accéder à une information détaillée sur ce qu'ils achètent, puis mangent, afin d'orienter notre agriculture par leurs choix de consommateurs. L'amendement n°

on fournirait une information qui, au-delà du score carbone d'un élevage, renseignerait l'acheteur sur le mode de production- au sol, avec un accès extérieur, en plein air, ou en agriculture biologique -afin de tenir compte de l'ensemble des enjeux de l'agroécologie et des attentes des consommateurs.

le consommateur sur les modes de production (utilisation ou non d'antibiotiques et d'activateurs de croissance, respect du bien-être animal, caractère transgénique des produits, » et de protéger les productions locales. Un tel étiquetage serait en outre conforme à la jurisprudence récente du Conseil d'État : la haute juridiction a jugé que les États membres peuvent imposer un étiquetage au nom de la protection des consommateurs s'ils attachent une importance significative à cette information et s'il existe un lien avéré entre certaines propriétés d'une denrée alimentaire et son origine ou sa provenance.

écologique), nous jetons chaque année 10 millions de tonnes de nourriture qui aurait pu être consommée. Ce gaspillage a bien évidemment un coût environnemental, mais il a également un coût économique : le gaspillage alimentaire représenterait en moyenne chaque année une perte de 100 euros par habitant.

pensant qu'il existe un danger sanitaire si un produit est consommé au-delà de la date de durabilité minimale, ce qui n'est bien évidemment pas le cas. Cette petite confusion est responsable de 20 % du gaspillage alimentaire des ménages.

indiquées sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire, en incitant à jeter des produits encore consommables. Sur un même produit, ces dates peuvent varier selon que celui-ci est commercialisé sur le territoire métropolitain ou outre-mer. Souvent, les dates limites sont repoussées outre-mer afin d'assurer la commercialisation

et d'améliorer l'information du consommateur quant à la possibilité de consommer ces produits au-delà de cette date. En effet, contrairement à la date limite de consommation, la date de durabilité minimale n'est qu'indicative, puisque le produit reste consommable sans entraîner de risques pour la santé.

accéder aisément à ces informations au moment de l'achat. Un affichage traditionnel peut être mis en place sans aucune complexité.

amendement, nous proposons de supprimer le renvoi au pouvoir réglementaire de la fixation des modalités d'application de l'article, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre.

Le calendrier de la saisonnalité des fruits et légumes change chaque année selon les aléas climatiques. Il faut également prendre en compte la question des variétés précoces et la pratique des légumes en primeur, afin de valoriser la production française face aux importations et de garantir la cohérence de notre action en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, il nous semble nécessaire d'associer les parties prenantes, à savoir la filière des fruits et légumes frais, à la détermination des modalités d'application de cet article. Tel est l'objet de cet amendement.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

à l'État de créer, éventuellement avec l'appui des collectivités territoriales concernées, des sociétés d'économie mixte dont l'objet unique serait l'aménagement et l'exploitation des terminaux multimodaux de fret.

groupe n'est pas favorable aux dispositions de cet amendement ; nous proposons, à l'inverse, un modèle économique qui s'appuie sur des ressources publiques pour moderniser les installations existantes, créer et financer les besoins nouveaux autour du gestionnaire du réseau, qui reste, aujourd'hui encore, la SNCF.

ces orientations, car nous considérons qu'il convient de laisser à l'État sa responsabilité en la matière, au travers des opérateurs publics, et de garantir l'unicité du réseau. Nous voterons donc contre cet amendement.

de la simple possibilité de prévoir, dans les conventions de terminal, la dégressivité d'une part du montant de la redevance due en fonction de la performance environnementale de la chaîne de transport. Il a ainsi pour objet de prévoir l'obligation d'introduire des clauses financières liées à des critères environnementaux, afin que des objectifs contractualisés de part modale, alliés à un signal prix tenant compte des externalités, soient mis en place par les ports.

de prévoir la dégressivité d'une part du montant de la redevance due en fonction de la performance environnementale de la chaîne de transport ainsi que l'instauration d'un objectif obligatoire de report modal seraient susceptibles d'entraîner une requalification des conventions de terminal en contrats de concession, puisque cela pourrait être assimilable

un outil prioritaire pour promouvoir la transition écologique et lutter contre la congestion routière, source de pollution et de nuisances importantes. La Convention citoyenne pour le climat a elle-même mis l'accent, dans son rapport, sur la nécessité de redonner une place plus

par wagon isolé, que nous proposons de déclarer d'intérêt général, au regard tant des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre que des enjeux d'aménagement du territoire. Les politiques libérales de réduction du réseau, de fermeture des gares et d'abandon de l'activité du wagon isolé ont conduit à mettre sur les routes des milliers de camions supplémentaires, ce qui est une ineptie. Nous ne sommes pas seuls à porter ces revendications. Ainsi, l'Association française du rail demande que le fret soit déclaré d'intérêt vital ; elle estime que, que, « dans la crise sans précédent que nous vivons, l'activité de fret ferroviaire est stratégique pour éviter une rupture dans la chaîne d'approvisionnement des entreprises. Le Gouvernement doit sans tarder adopter des mesures concrètes de sauvegarde en faveur des entreprises engagées dans le fret ferroviaire, pour assurer la continuité du service. »

de cette stratégie. Il semble par conséquent plus opportun de faire du développement du wagon isolé, outil particulièrement pertinent à l'heure où nos flux sont de plus en plus éclatés, une part intégrante de cette stratégie.

Pour que les investissements soient efficaces et efficients, il est nécessaire que la stratégie prenne en compte concrètement l'organisation industrielle dans les territoires, le futur des biens à transporter, les niveaux de service exigés par les commanditaires

l'octroi des permis et autorisations de réalisation ou d'agrandissement des plateformes logistiques à la présentation

ont pu montrer les limites du recours à ce critère dans le cadre de politiques environnementales et climatiques. En effet, il s'agit d'un indicateur imparfait de l'impact climatique des poids lourds.

que l'État assure un suivi de la formation à l'écoconduite des chauffeurs routiers. Le potentiel est important. En effet, si l'écoconduite devenait la pratique courante, elle pourrait permettre, nous dit-on, une réduction de 15 % de la consommation de carburant des poids lourds. Quel est l'avis de L'article 31 inclut déjà l'écoconduite dans la formation initiale et continue des conducteurs de poids lourds sans en modifier sensiblement la charge pour les entreprises,

Dans le souci de ne pas alourdir les dispositifs pour les entreprises, nous proposons par cet amendement d'inscrire la réduction de l'incidence de la conduite des conducteurs routiers sur l'environnement dans le cadre de leur qualification initiale et des sessions de formation continue, d'une durée de cinq jours, renouvelables tous les cinq

Merci

ou de carte grise. L'absence de régulation de ces plateformes comporte des risques pour la sécurité routière et la sécurité sociale, mais également pour la préservation de l'environnement. Le présent amendement vise donc à créer une nouvelle obligation pour les opérateurs de plateformes numériques, afin qu'ils s'assurent de la bonne connaissance des pratiques d'écoconduite et des règles de sécurité parmi les conducteurs ayant recours à leur service.

soulève d'ailleurs de nombreuses questions relatives au statut des travailleurs. Par ailleurs, aucun mécanisme de contrôle ou de sanction n'est prévu, ce qui réduirait certainement son applicabilité. La commission a donc émis un avis défavorable sur

Les formations de sensibilisation à l'écoconduite qui figurent à l'article 31 constituent des contraintes humaines, matérielles et financières pour les entreprises et les collectivités. Cet amendement a donc pour objet de le supprimer.